En effet, elles redoutent notamment que la généralisation de la déclaration sociale nominative à tous les employeurs, prévue à l'alinéa 3, ne puisse être remise en cause par l'alinéa suivant, qui indique que les dispositions du chapitre en question qu'aux entreprises de plus de 20 salariés. Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement l'obligation déclarative, élargie à tous les employeurs. C'est une très bonne mesure, car elle permettra de dresser une cartographie précise de l'emploi des personnes en situation de handicap.

En effet, elle limite la mesure aux entreprises de plus de 250 salariés. Le rapporteur prétextera qu'il s'agit de protéger les TPE-PME. néanmoins que les TPE ne sont pas concernées par l'OETH, qui ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 20 salariés. Par ailleurs, il paraît opportun que, pour une entreprise à établissements multiples, l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'effectue à l'échelon de l'entreprise et non plus de l'établissement. En effet, aujourd'hui, dans le secteur privé, l'assujettissement à cette obligation est réalisé au niveau de l'établissement autonome, une notion qui n'existe pour aucune autre contribution. Cette modification permettrait donc à la fois de simplifier les formalités de l'entreprise et d'éviter les risques d'éviction lorsqu'une entreprise compte de compte de multiples petits établissements. Monsieur le rapporteur, Il est en effet apparu que l'idée du Gouvernement d'appliquer l'OETH à l'échelon de l'entreprise et non plus de l'établissement n'était sans doute pas compatible avec un modèle économique construit autour de l'éclatement de petites entités. le présent amendement, il est suggéré de maintenir le calcul établissement par établissement, à la condition de la signature d'un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d'entreprise, dont le dispositif renvoie à un autre amendement, que je défendrai plus tard. À défaut de cette signature, le principe de l'acquittement au niveau de l'entreprise s'appliquerait.

Apourceau-Poly. L'article 40 redéfinit l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans le secteur privé ou public pour tout établissement d'au moins 20 salariés.

les entreprises pouvaient comptabiliser les sociétés de sous-traitance employant des personnes en situation de handicap et compter les élèves handicapés en stage en leur sein. Sous couvert de simplification de la déclaration et du nombre de travailleurs handicapés, le Gouvernement exonère toujours plus les entreprises de leurs obligations. Ainsi, les dépenses destinées à favoriser l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés pourront être déduites de la contribution versée par les entreprises qui ne disposent pas de 6 % de travailleurs handicapés. Autrement dit, ce sont les personnes en situation de handicap qui financent elles-mêmes les travaux d'adaptation dans les entreprises que les patrons refusent de financer eux-mêmes. L'assouplissement des obligations en matière d'emploi des employeurs publics et privés ne pourrait s'entendre que si l'objectif de 6 % était atteint dans les établissements et si le taux de chômage des personnes en situation de handicap n'était pas de 19 %, soit près de deux fois de deux fois supérieur au taux moyen de chômage de la population. Nous ne pensons pas que le fait de développer l'emploi précaire en intérim sera de nature à répondre aux exigences d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Si, aujourd'hui, les entreprises sont réticentes à adapter leurs locaux aux personnes en situation de handicap, il paraît peu crédible que les sociétés d'intérim réalisent des travaux pour ces travailleurs dont la situation est plus qu'incertaine.

encore de prêt-à-porter pourraient ainsi facilement être exonérées de l'OETH. Cet amendement tend donc à abaisser ce seuil à 50 salariés, afin de conserver une réelle ambition pour l'obligation d'emploi. Grelet-Certenais. Cet amendement vise à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 5212-7 du code du travail, car les modifications proposées par le présent projet de loi constituent une atteinte aux principes mêmes de l'OETH.

à 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. Si l'accès aux stages ou à l'immersion représente effectivement l'une des voies pour massifier l'emploi des personnes en situation de handicap, cette possibilité figure déjà dans la loi et permet aux employeurs d'intégrer ces types d'emploi dans le calcul du quota. En supprimant le plafond de recours aux stages et autres, le risque existe de fragiliser et de dénaturer ainsi l'OETH. L'emploi, y compris pour les personnes en situation de handicap, c'est avant tout un véritable contrat de travail.

qui tend à conserver le dispositif proposé par le Gouvernement, tout en posant deux garde-fous essentiels pour préserver l'ambition première de l'obligation d'emploi. Nous proposons donc de réaffirmer que le recours aux stages ou aux immersions pour satisfaire les exigences de l'OETH ne peut être que partiel,

Monsieur le rapporteur, est une préoccupation majeure qui reste cependant trop souvent oubliée. L'article 40, qui a précisément pour objet de valoriser l'emploi des travailleurs handicapés seniors, mériterait d'être réécrit, afin de gagner en intelligibilité et en cohérence, au regard des principes qui doivent être posés dans la loi sur ce sujet, notamment les modalités précises de mise en oeuvre, qui relèvent bien du domaine réglementaire.

Les délais de mise en oeuvre envisagés par le Gouvernement, et définis par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale, sont trop longs au regard des objectifs de la réforme- c'est ce que nous ont dit de nombreuses associations. C'est pourquoi cet amendement tend à une accélération de la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi pour les entreprises à établissements multiples.

cet amendement. L'amendement n° 492 vise à supprimer l'ensemble des modalités introduites par le Gouvernement pour favoriser l'emploi direct des personnes handicapées, notamment le changement de périmètre de déduction des montants des contrats de sous-traitance avec les ESAT et les entreprises adaptées. En effet, le projet de loi entend déduire ces montants du niveau non plus de l'obligation, mais de la contribution financière dont sont redevables les entreprises qui ne comprendront pas 6 % de salariés handicapés. Cette nouvelle forme de déduction a pour objet de réduire la mise en oeuvre indirecte de l'obligation par des recours à des contrats externes, et de favoriser l'emploi direct. Nous ne pouvons que nous montrer défavorables à cet amendement, car il remet en cause l'esprit du texte que nous soutenons.

à l'amendement n° 389, en raison de la volonté très claire exprimée par les associations de travailleurs handicapés elles-mêmes de réduire toute forme d'entrave possible à l'embauche. Toutes les formes d'emploi, englobant même les stages et les emplois intérimaires, doivent être ouvertes sans restriction aux travailleurs handicapés.

La rédaction de l'amendement n° 634 n'est satisfaisante qu'en apparence : celui-ci tend, certes, à revenir sur la position du Gouvernement qui limitait la possibilité pour les employeurs de moduler leur contribution en fonction des seuls bénéficiaires de l'obligation ayant un certain âge. la disposition retenue revenait entièrement sur le droit en vigueur, qui prévoit la même modulation pour les bénéficiaires dont le handicap est particulièrement lourd, pour ceux qui sont en chômage de longue durée ou pour ceux qui viennent d'ESAT ou d'entreprise adaptée. Elle était donc contraire à l'objectif d'inclusion des travailleurs handicapés les plus éloignés de l'emploi. La nouvelle rédaction suggérée par les auteurs de cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l'âge des bénéficiaires, pour revenir à la notion plus large de « difficultés particulières », ce qui semble aller dans le bon sens. Pour autant, son objet vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés seniors. Est donc réaffirmée, implicitement, la volonté du Gouvernement de réserver les seuls critères de modulation de la contribution aux bénéficiaires âgés. Or nous souhaitons que les autres critères actuels soient également maintenus.

n° 633 tend à assujettir toutes les entreprises à établissements multiples au niveau de l'entreprise en supprimant le seuil de 250 salariés introduit par la commission des affaires sociales du Sénat. Je suis favorable à cet amendement, qui est conforme à l'esprit et à la lettre de la réforme de l'obligation d'emploi telle qu'elle a été présentée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale. L'assujettissement à l'échelon de l'entreprise permet de simplifier les formalités des entreprises ; il est cohérent avec le niveau de pilotage des politiques des ressources humaines. Afin de maîtriser l'effet de cette mesure sur les charges des entreprises, il est prévu d'encadrer de façon provisoire les éventuelles augmentations de la contribution qu'une entreprise assujettie serait amenée à supporter. Le Gouvernement est en revanche

Le scrutin est ouvert.

En effet, ce sont ces derniers qui font le choix de rejoindre une telle entreprise. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l'intégration de personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage. Quel est l'avis de commission ? Juridiquement, les modèles économiques de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise de portage salarial sont assez proches : les deux reposent en effet sur la mise à disposition lucrative d'une partie de leurs salariés. Or la loi prévoit que les entreprises de travail temporaire ne sont redevables de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés que pour la part permanente de leurs salariés, admettant donc le principe d'une OETH au périmètre réduit. En toute logique, le même principe devrait s'appliquer aux entreprises de portage salarial. La commission émet donc un avis favorable

salariés portés. Mais cette mesure relative au décompte des effectifs des entreprises mérite une expertise complémentaire et pourrait être examinée dans le cadre du projet de loi PACTE, ou plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dont certaines dispositions portent précisément sur cette thématique. C'est pourquoi le Gouvernement

n° 414 rectifié . L'article 40 prévoit la fin des accords dits « agréés », en limitant leur durée à six ans maximum. Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas été invités à participer à la concertation Or celui-ci aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions « handicap » des établissements d'enseignement supérieur, tant privés que publics.

Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés- il s'agit du soutien à la formation des personnes handicapées et du -qui leur permettent d'accompagner au mieux les étudiants, avec une vision à long terme. La fin des accords agréés affecterait directement et durablement l'accès à l'enseignement supérieur des personnes en situation de handicap et, partant, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer ni les aménagements, qu'il s'agisse du mobilier, du matériel ou des aides humaines, ni les frais annexes- assurances, surcoûts discriminatoires, etc. Cet amendement vise donc à supprimer la limitation dans le temps des accords agréés,

M. Martin Lévrier. L'article 40 dispose que l'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé comprenant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de cumuler l'aide financière apportée à l'embauche par l'AGEFIPH et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée. À nos yeux, ces deux mécanismes d'incitation financière peuvent servir des objectifs différents : le maintien dans l'emploi pour le premier, l'embauche pour le second. La règle de leur non-cumul ne répond donc pas à un impératif d'efficacité ou d'économie. Elle doit, dès lors, être

ne s'applique pas spécifiquement à une catégorie de travailleurs. La mesure que vous proposez n'aurait donc pas d'effet concret. Surtout, le télétravail est une forme d'organisation qui implique une réflexion quant aux méthodes et aux structures de production de l'entreprise. Il doit donc demeurer un outil concerté entre le salarié et son employeur. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à déployer un plan global d'aide aux aidants. Ce plan comprendra un volet relatif à l'amélioration des conditions de l'articulation entre vie professionnelle et soutien aux personnes âgées. Des mesures seront donc rapidement prises dans ce cadre. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

permettent notamment d'éviter les déplacements du domicile au lieu de travail : dont acte. Toutefois, il nous semble essentiel de compléter cet article, afin d'encadrer le recours au télétravail pour les personnes en situation de handicap. À travers cet amendement, nous soulevons deux enjeux distincts.

à ses devoirs. De fait, en encadrant le télétravail des personnes en situation de handicap, particulièrement en prévoyant que ces télétravailleurs ou télétravailleuses sont appelés à se présenter dans l'entreprise régulièrement et qu'ils y disposent de locaux, on reste dans l'esprit de l'article

En effet, tel que l'article 40 est rédigé, c'est un véritable régime dérogatoire qui est prévu, lequel risque de conduire à l'isolement de personnes qui ne demandent qu'à être intégrées dans une équipe. L'enjeu est donc bien d'assurer une insertion adaptée dans l'entreprise, ce qui doit passer par un minimum de présence dans les locaux, avec les collègues. Ce faisant, on permet de créer des liens conduisant, d'ailleurs, à une meilleure synergie des équipes.

vous proposez ne sont pas cohérentes avec la nouvelle architecture conventionnelle issue des ordonnances Travail adoptées à l'automne dernier. Désormais, la négociation obligatoire porte sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

cet amendement vise à transposer, dans notre législation nationale relative aux discriminations fondées sur le handicap, l'obligation d'aménagement raisonnable définie par l'article 5 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

L'article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH, ratifiée par la France en 2010, mentionne : « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable ». Cet amendement tend donc à pallier le caractère insuffisant de notre législation, afin de sécuriser le droit national et d'améliorer les conditions d'accès et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap.

cet article, « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement [ ...] de son handicap [ ...], une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ». En outre, la discrimination indirecte est définie comme la disposition susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres. Or le Or le défaut d'aménagement du poste de travail par l'employeur, en ce qu'il place la personne handicapée dans une situation moins favorable ou entraîne pour elle un désavantage particulier, est déjà parfaitement constitutif d'une discrimination directe ou indirecte. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

La commission avait souhaité accompagner le mouvement, engagé par le Gouvernement, de rapprochement des modalités de calcul de l'obligation en question dans les secteurs privé et public, en retirant les agents reclassés des bénéficiaires de l'obligation.

le rapporteur. Avec cet amendement, nous nous penchons sur le cas particulier de certains corps spécialisés de la fonction publique, dont l'accès est régi par des conditions d'aptitudes physiques singulières. Je pense notamment aux services départementaux d'incendie et de secours,

les critères d'aptitude physique ou d'âge, évoqués par M. le rapporteur, peuvent trouver une forme d'application dans le secteur privé, mais n'ont jamais été appliqués dans le secteur public. Aussi, nous considérons que l'adoption de cet amendement aurait pour effet de restreindre le champ d'application des règles d'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable.

secrétaire d'État. Dans le cadre de la réforme en cours, le Gouvernement souhaite que les efforts réalisés par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes lourdement handicapées n'entraînent plus une majoration du taux d'emploi.

les écoles et les universités, avec, pour ces dernières, un plafonnement de la déduction à 80 % de la contribution exigible en 2006 et à 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement devait être revu annuellement : mais la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé ce plafonnement. Le plafonnement

Au regard de la massification des dispositifs de prise en charge des élèves handicapés observée au cours des dernières années, cette évolution fiabilise le mécanisme proposé et justifie un abaissement substantiel du taux de plafonnement. Avec cet amendement, nous réaffirmons donc le principe d'exemplarité des pouvoirs publics, notamment de l'éducation nationale.

Apourceau-Poly. L'emploi des personnes en situation de handicap doit être une priorité partagée par toutes et tous. En pratique, pourtant, la contribution acquittée en cas de non-respect de l'obligation de recrutement fait autant figure de sanction que d'une option visant à permettre ce recrutement. Dans ce cadre, il me semble déjà problématique que les établissements scolaires puissent déduire de leur contribution les salaires des personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap, pour deux raisons.

et tous à l'instruction. De fait, si ces personnels d'accompagnement planifiés dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation sont indispensables, ils répondent à une exigence fixée par la loi. Toutefois, il faut bien reconnaître aujourd'hui, il est difficile pour les établissements de faire face à la pénurie budgétaire qui touche tous les secteurs de l'État. Dans ce contexte, la déduction des charges est non pas un cadeau, mais une nécessité.

les réponses restent insuffisantes, notamment en ce qui concerne le temps périscolaire. Malgré les préconisations formulées par le Défenseur des droits dès 2012 et malgré la jurisprudence du Conseil d'État du 20 avril 2011, on ne peut pas dire que l'État ait mis en oeuvre les moyens suffisants pour permettre l'accès des enfants en situation de handicap aux temps scolaires et périscolaires. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont conduit à l'augmentation drastique des inscriptions scolaires d'enfants français en situation de handicap

Jusqu'à l'année en cours, les montants de masse salariale affectés à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap dans les écoles étaient déduits de la contribution versée par l'employeur éducation nationale au FIPHFP.

je crois que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose. Le Gouvernement ne propose pas de minorer le montant des rémunérations prises en compte pour calculer le montant de la contribution. Il souhaite que, quel que soit le montant des rémunérations consacrées

afin de sécuriser financièrement ces structures spécifiques, qui ont besoin de visibilité et, surtout, de continuité budgétaire pour assurer leurs missions.

de la commission ? La commission s'est montrée attentive à ce que l'instrument contractuel signé par l'entreprise adaptée et l'autorité d'agrément ne soit pas de même nature que ceux qui ont cours dans le milieu médico-social. Il ne s'agit pas pour nous de nier la dimension financière des relations entre l'État et les entreprises adaptées, qui font d'ailleurs l'objet de modifications importantes. Mais nous tenions à rappeler que le subventionnement des entreprises adaptées

Il me paraît important que la question des moyens soit réintégrée dans l'intitulé du nouvel outil contractuel qui liera les entreprises adaptées et l'État. Le principe d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est

Le dispositif adopté par la commission tend à donner des objectifs aux entreprises adaptées pour qu'elles conduisent les personnes qu'elles font travailler vers l'emploi durable. Or, pour de nombreuses personnes en situation de handicap,

Les amendements déposés par le Gouvernement allant dans le sens d'une plus grande porosité entre entreprises adaptées et entreprises dites classiques vont d'ailleurs implicitement dans ce sens. Les auteurs de l'amendement n° 393 souhaitent que soit gommée toute mention dans la loi d'une non-appartenance des entreprises adaptées

de l'évolution que vous avez bien comprise et qui va dans le sens de ce que nous souhaitons et que souhaite le secteur des entreprises adaptées : ces entreprises ne fournissent pas seulement un travail à des personnes en situation de handicap ; elles permettent à tous ceux qui le peuvent d'aller vers

à Pôle emploi et n'arrivent pas à accéder au marché du travail. Notre objectif est de doubler d'ici à quatre ans le nombre de personnes susceptibles de travailler en entreprise adaptée,

Les quatre amendements que le Gouvernement a déposés traduisent cette volonté partagée de transformation, sans renier les réalités et les spécificités des entreprises adaptées, qui jouent un rôle essentiel dans notre pays.

Enfin, de concert avec Nicole Belloubet, il vous sera proposé de renforcer les chances de réinsertion sociale et professionnelle des détenus en offrant à ces derniers des activités au sein d'entreprises adaptées.

de rationaliser l'aide financière au poste et de la réserver aux travailleurs handicapés. La disparition de la subvention spécifique dont bénéficiaient les entreprises adaptées au profit de l'aide au poste est sans doute une mesure de bonne gestion. Ensuite, il est proposé que, si un salarié d'une entreprise adaptée souhaite intégrer une autre entreprise, cette dernière bénéficie d'un appui individualisé à l'intégration du salarié.

courent le risque de perdre leur emploi ». Cette proposition ne me semble pas réalisable, dans la mesure où l'aide financière n'est versée qu'à raison des travailleurs effectivement embauchés par les entreprises adaptées, donc nécessairement titulaires d'un emploi. Je propose aux auteurs de cet amendement de se rallier à celui du Gouvernement qui vise à limiter l'aide financière au poste aux travailleurs handicapés en entreprise

nous partageons l'objectif d'une véritable chaîne d'accès à l'emploi pour une société plus inclusive, mais pas de cette manière. Vous nous demandez de nous prononcer sur cette évolution majeure sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Madame la ministre, vous savez pourtant comment les groupes politiques travaillent en amont de l'examen en séance des projets de loi. Mon groupe a auditionné de nombreux acteurs du secteur de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais nous n'avons évidemment pas été en mesure de les consulter sur l'évolution majeure Je regrette que votre gestion de la réforme par à-coups nous empêche d'appréhender et, surtout, d'apprécier les changements dans leur globalité. Ce n'est assurément pas de bonne méthode ! Cette évolution nous inspire à tout le moins de fortes questions. De fait, nous ne partageons pas la même philosophie : pour nous, les entreprises adaptées ne sont pas un tremplin vers le milieu ordinaire ; elles sont une facette de ce milieu très

par exemple, les accidentés du travail avec incapacité permanente, les victimes de guerre, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou les attributaires de l'allocation

Elles sont donc considérées comme les usagers d'un établissement social et signent à ce titre un contrat de soutien et d'aide par le travail prévu par le code de l'action sociale et des familles. Il n'est pas possible juridiquement d'ouvrir à ces personnes des droits à l'assurance chômage sans remettre

En effet, l'intégralité des dispositifs qui s'appliquent aux entreprises adaptées, notamment les aides financières dont elles peuvent bénéficier à l'embauche d'un travailleur handicapé, est conditionnée, d'après le nouvel article L. 5213-13-1 du code du travail, à la signature d'un contrat de travail entre l'entreprise et le travailleur. Or le travail de la personne détenue est encadré par un acte spécifique, dont ne sont signataires que la personne et le chef d'établissement pénitentiaire, et qui n'a pas la qualification de contrat de travail. L'incitation de l'entreprise adaptée à solliciter le travail d'une personne handicapée détenue, qui n'est pas couverte par un contrat de travail et n'ouvre le droit à aucune aide, me paraît donc fortement diminuée. Je crains que le dispositif proposé ne trouve pas d'effectivité. La commission s'en remet donc à la sagesse

? Cet amendement complète utilement l'ensemble des mesures prises en commission des affaires sociales et destinées à protéger les parcours qui vont vers plus d'autonomisation et plus de protection. Pour mémoire, la commission s'était surtout attachée à sécuriser les parcours qui vont vers plus d'autonomisation, derniers concernant les travailleurs d'ESAT désireux d'intégrer le milieu adapté ou le milieu classique de travail. L'article additionnel que le Gouvernement propose d'introduire concerne les parcours qui vont vers plus de protection, en permettant à des travailleurs handicapés sans emploi ou menacés par une perte d'emploi de signer un CDD de quatre à vingt-quatre mois avec une entreprise adaptée, laquelle disposera pour ce faire des aides financières attribuées

Nadine Grelet-Certenais. La réécriture de l'article 47 de la loi de 2005 proposée par le Gouvernement supprime la référence aux normes internationales en matière d'accessibilité, référence maintenue dans la récente loi pour une République numérique. Cette évolution implique que les seules références à des normes d'accessibilité seraient donc celles qui sont inscrites dans le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, le RGAA. En raison du contexte numérique international et de l'importance du réseau mondial francophone,

que le référentiel général pour l'accessibilité des administrations mentionné dans l'objet de l'amendement est parfaitement à jour des recommandations internationales et continuera de s'appliquer en tenant compte de la charge disproportionnée qu'induira l'accessibilité numérique d'un service.

Elle permet l'acquisition de compétences et de qualifications correspondant aux besoins du marché du travail et au projet professionnel de la personne. Cet amendement tend à modifier la définition législative du secteur de l'insertion par l'activité économique dans le code du travail. Il s'agit de faire apparaître officiellement cette mission de formation professionnelle et de traduire dans la loi le triptyque « mise à l'emploi, accompagnement, formation

l'amendement n° 397. Cet amendement vise à modifier la définition législative de l'insertion par l'activité économique dans le code du travail en y incorporant la mission de formation. L'insertion par l'activité économique, ou IAE, permet avant tout aux personnes les plus éloignées de l'emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle.

les bénéficiaires de l'IAE sont également formés au sein de structures spécialisées telles que les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d'insertion ou les ateliers et chantiers d'insertion. Cela contribue fortement à l'innovation sociale au service de la lutte contre les exclusions du marché du travail. Par ailleurs, l'inclusion dans l'emploi ne relève pas de la seule responsabilité des chômeurs, bien au contraire. C'est une responsabilité partagée qui doit passer par un changement du regard porté sur le demandeur d'emploi, une sortie des préjugés en quelque sorte, parfois par un engagement de l'employeur.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l'État de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l'emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l'État y donne suite, ce qui témoigne des limites de l'outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L'expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l'emploi, alors que dans le cadre d'une délégation de compétence, elles agissent au nom et pour le compte de l'État.

que l'article 7 de la loi NOTRe a vu le jour, dans une version certes moins ambitieuse que ce que souhaitait le Sénat. Ensuite, la loi NOTRe ne prévoit pas un transfert de compétence, mais une délégation de pouvoir aux régions pour qu'elles agissent au nom de l'État, ce qui n'est pas du tout la même chose. En outre, le passage à une expérimentation n'apporte aucune garantie à l'État par rapport au droit en vigueur, car dans les deux cas tout dépendra de la volonté de l'État de confier aux régions de nouvelles missions. Par ailleurs, l'expérimentation proposée prévoit que les régions coordonnent l'action de tous les acteurs de la politique de l'emploi, y compris Pôle emploi. Enfin et surtout, le Sénat a adopté le 13 juin dernier la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale présentée par nos collègues Bruno Retailleau et Philippe Bas, qui modifie également les compétences des régions en matière d'emploi.

un dispositif ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi qui ont des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce dispositif permettrait ainsi à des collectivités territoriales d'embaucher en CDD d'insertion des personnes éloignées de l'emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d'une entreprise. Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer progressivement le monde du travail. Il s'agit ainsi, au travers de cet outil, de multiplier les occasions de contacts entre les personnes en insertion et le monde de l'entreprise tout en permettant aux collectivités volontaires- exclusivement volontaires -, de s'investir davantage dans l'activation des dépenses passives et l'inclusion dans l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Quel est l'avis de la commission ? Nous avons

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, le secteur du bâtiment a connu depuis 2004, mais surtout depuis 2012 avec la crise économique des pays du sud de l'Europe, un développement considérable du travail détaché. En 2017, le BTP représentait le troisième secteur en termes de déclarations de détachement et de nombre de salariés détachés. Face à ce phénomène massif, l'enjeu principal est la lutte contre la fraude au détachement à l'origine d'une concurrence sociale déloyale qui pénalise sévèrement les entreprises et l'emploi. Si les professionnels sont favorables au développement du marché européen, il importe cependant qu'il se développe dans des conditions de concurrence sociale loyales. Sans même évoquer les salaires indignes, la fraude se caractérise souvent par une fraude aux horaires ou sur le niveau du salaire versé. Ainsi, les prix pratiqués par les entreprises sont tellement tirés vers le bas qu'il est impossible pour les entreprises établies sur notre territoire national de les concurrencer. Ces dernières années, la lutte contre les fraudes au détachement a fait l'objet de nombreuses dispositions, mais la mobilisation des services de contrôle reste encore insuffisante. Les sanctions administratives en matière de fraude au détachement et de travail illégal prévues à l'article 53 permettent la mise en oeuvre d'un arsenal répressif complet, grâce notamment à l'extension de la définition du travail dissimulé au cas des sociétés boîtes aux lettres. En revanche, concernant le devoir de vigilance des maîtres d'ouvrage à l'égard des cocontractants prévu à l'article 54, si la recherche de l'effectivité des sanctions est un objectif louable d'un point de vue de vue opérationnel, nous pouvons nous interroger sur la mise en oeuvre pratique d'un tel dispositif. Je terminerai en insistant sur la vigilance accrue qu'il conviendra également d'exercer concernant les travailleurs étrangers qui, employés dans des exploitations agricoles françaises, bénéficient des allocations de l'assurance chômage une fois rentrés chez eux et exercent une nouvelle activité dans leur pays d'origine pour obtenir, dans un second temps, de nouvelles allocations.

parmi lesquels 75 000 Portugais, 60 000 Polonais, 45 000 Allemands et quasiment autant de Roumains. C'est un flux qualifié, qui complète de manière parfois spectaculaire l'immigration respective de chacun de ces pays en France et montre le caractère qu'il convient de donner au détachement, détachement, celui d'une gestion des ressources humaines permettant de contourner habilement une bonne partie des obligations que les employeurs doivent remplir au regard de la loi. C'est aussi une bonne manière de conjuguer, notamment, construction européenne et moins-disant social. De notre point de vue, le jeu sur les différentiels sociaux est, somme toute, relativement secondaire : ce qui est en jeu est bien plutôt, en l'espèce, une façon comme une autre de gérer au mieux les coûts par le recours à la sous-traitance,

qui tend, en même temps, à renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail dans ses contrôles et ses sanctions contre la fraude au travail détaché et à alléger les obligations pesant sur les employeurs qui y ont recours. Par ailleurs, le cadre législatif du travail détaché est remanié tellement régulièrement que l'inspection du travail n'a pas le temps d'intégrer ces modifications que ces dernières ont déjà changé. En outre, une nouvelle directive européenne vient d'être adoptée en ce domaine, comme mon collègue l'a souligné. Inutile donc de modifier une énième fois le dispositif avant la transposition de ladite directive.

nous le savons, on enregistre une baisse continue du nombre d'agents de contrôle, qu'ils soient contrôleurs du travail ou inspecteurs du travail.

vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de problème, puisque le nombre d'inspecteurs ou d'agents de contrôle était suffisant au regard des normes de l'Organisation internationale du travail et que, surtout, vous aviez recentré les priorités de l'inspection du travail

transfrontalières. Résidant sur un territoire transfrontalier franco-luxembourgeois, à un kilomètre de la frontière, je constate que les frontières sont abolies par un espace de vie en commun. Des espaces contigus ou, en tout cas, de coopération existent

Cohen, pour présenter l'amendement n° 227 Il fallait faire évoluer la législation sur le travail détaché en permettant, notamment, aux entreprises étrangères sans représentation dans notre pays de détacher temporairement un ou plusieurs salariés, en vue d'y réaliser, par exemple, une mission commerciale ponctuelle. En l'espèce, l'entreprise n'aurait plus l'obligation de déclaration par le biais d'un correspondant et devrait en quelque sorte se débrouiller toute seule avec l'inspection du travail en France. Cela va nécessiter une très forte mobilisation

M. Fabien Gay. Dans les faits, le code actuel fixait une contribution minimale des entreprises étrangères pour faciliter la mise en place du système de traitement des données. Il faut croire que les moyens de conception et de mise en oeuvre de ce système ont été réunis, puisque l'article 52 prévoit la suppression pure et simple de la contribution. À la vérité, la contribution n'a jamais fait l'objet du moindre recouvrement, alors même que, comme beaucoup d'impôts de faible quotité, elle présentait l'avantage de permettre l'identification des entreprises recourant au travail détaché. On notera que, en même temps, pour tenir l'équilibre, d'une certaine manière, l'article 53 prévoit de majorer les amendes administratives pour infraction au travail détaché, sans en majorer le montant maximal, soit dit en passant. Pour notre part, nous préférons tirer parti de la discussion de ce projet de loi pour modifier le contenu de cet article du code du travail. En lieu et place d'un financement des systèmes d'information du ministère du travail, qui n'a d'ailleurs jamais été mis en place nous sommes partisans du versement d'une sorte de différentiel des cotisations sociales patronales, au bénéfice de notre système de sécurité sociale. Les modes de financement de la sécurité sociale sont différents d'un pays l'autre et les taux applicables aux cotisations de la part patronale plutôt variables. Seuls, en effet, les deux royaumes de Suède et de Belgique ont des montants de cotisations patronales plus élevés. Mais il convient de noter que, si les coûts du travail dans l'industrie sont proches en France et en Allemagne, l'Allemagne dispose d'un différentiel en sa faveur dans le secteur des services, fondé sur le développement d'un grand nombre de « petits boulots » mal payés dans le domaine des services connexes aux activités industrielles. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'on a créé en France le CICE, et mis en oeuvre le pacte de responsabilité et de solidarité. Objectif dépassé au-delà de toute espérance : 29 % des contrats de travail signés depuis le début de l'année sont des contrats d'un jour ! Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter,

prévoit que ce sont les règles du pays d'origine qui s'appliquent pendant les deux premières années d'un détachement en matière de sécurité sociale. J'ajoute que la Commission européenne a présenté en décembre 2016 une proposition de révision de ce règlement, qui est toujours débattue. Aussi, je vous invite à y apporter votre contribution. Avec vous ! En tout état de cause, la commission est défavorable

suffisamment importante pour justifier, sinon un débat sur la transposition de la directive dans le présent texte, à tout le moins le dépôt d'un texte en bonne et due forme, une fois les travaux nécessaires accomplis. En matière de travail détaché, nous avons souligné le fait que plus de 500 000

Polonais, les Allemands et les Roumains, les Français détachés en France venant en cinquième position. Le « top 5 » des déclarants, si je puis m'exprimer ainsi, place dans l'ordre : l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie. La Pologne vient ensuite, avec environ quatre fois moins de salariés déclarés par des entreprises polonaises que de salariés détachés, suivie du Luxembourg qui, apparemment, compte un certain nombre de donneurs d'ordre. Dans les pays récemment entrés dans l'Union européenne, l'émigration des travailleurs et le travail détaché agissent comme des soupapes de sécurité pour fluidifier le marché du travail local, en relâchant la pression sur la demande d'emploi. Il faut d'ailleurs reconnaître que la France elle-même est déjà confrontée au phénomène, qu'il s'agisse de la Lorraine à proximité du Grand-Duché du Luxembourg, grand pourvoyeur d'emplois industriels, commerciaux et bancaires pour les pays voisins, ou de cette même région et de l'Alsace vis-à-vis de l'Allemagne, sans parler de l'attractivité de la République de Genève sur les habitants de la Haute-Savoie. On rappellera ici que près de 900 000 jeunes de 25 à 34 ans, formés dans les écoles, les lycées, les centres d'apprentissage et les universités françaises, font le bonheur des économies étrangères où ils ont pu faire valoir leurs diplômes et leurs talents. Le moins-disant social étant puissamment à l'oeuvre à l'échelon européen, seule une discussion parlementaire

à mettre un terme à la concurrence déloyale, au social et, enfin, à imposer des conditions de travail équitables, ainsi qu'une règle commune simple : à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail Nous regrettons toutefois que le Gouvernement n'ait pas estimé suffisamment important d'aller jusqu'au bout de la démarche engagée avec cette directive, en en faisant un texte de portée universelle pour tous les travailleurs, y compris les transporteurs routiers.

il est difficile aujourd'hui d'obtenir de telles garanties en dehors de la directive. Dans la négociation du paquet Mobilité au Parlement européen, la droite européenne n'a ainsi pas hésité à remettre à plat tous leurs droits et à contester pied à pied toutes les avancées négociées l'an dernier, qui auraient pu être intégrées à la directive relative au détachement des travailleurs. travailleurs. Madame la ministre, nous estimons que ce texte si important mérite mieux qu'une transposition par voie d'ordonnance : la révision de cette directive, qui conforte des droits concrets pour nos concitoyens, qui porte une vision sociale et qui démontre que l'Europe peut peut répondre présent, lorsqu'il s'agit de mieux les protéger, devrait faire l'objet d'un projet de loi ordinaire, avec un débat qui permettrait d'apporter une image plus positive et plus concrète de l'Europe, notamment dans la perspective des prochaines élections européennes. Pour ces raisons, nous voterons contre votre amendement.

Je n'ai strictement rien contre les frontaliers qui trouvent des accords de part et d'autre de la frontière : cela me paraît parfaitement logique. Je n'ai rien non plus contre les travailleurs d'autres pays européens qui viennent remplir une mission que l'on ne peut pas remplir nous-mêmes.

Aujourd'hui, on recourt de plus en plus à des plateformes- c'est le nouveau mot à la mode -, qui sont situées un peu partout, et qui effectuent toutes les formalités nécessaires pour amener dans nos territoires des travailleurs qui sont réputés en règle.

Requier, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié. Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation à la charge des donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, qui consiste à vérifier, lors de la conclusion du contrat, que le cocontractant s'est acquitté du paiement d'éventuelles amendes prononcées par l'administration à son encontre. Les donneurs d'ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l'égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs, et parfois indirects : vigilance sur le travail dissimulé, sur l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, sur l'agrément des sous-traitants ... Cette nouvelle obligation soulève des questions. Comment vérifier, en pratique, que le cocontractant a bien payé les amendes dont il était redevable ? Le projet de loi est silencieux sur les modalités de cette vérification. Une attestation sur l'honneur sera-t-elle suffisante ? Rappelons que la déclaration subsidiaire que le donneur d'ordre est tenu d'effectuer, en l'absence de déclaration préalable de détachement effectuée par son cocontractant, n'est applicable que lorsque ce dernier est lui-même tenu d'effectuer une telle déclaration préalable. En outre, les entreprises effectuant des prestations de courte durée, listées par l'arrêté qui devrait prochainement paraître, ne seront pas tenues d'effectuer une déclaration préalable de détachement. Rien dans la rédaction actuelle du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ne permet d'écarter avec certitude l'obligation de déclaration subsidiaire dans une telle hypothèse.

les modalités de mise en oeuvre de la procédure de suspension doivent être précisées. Il est déjà prévu qu'elles le soient dans un décret en Conseil d'État. Les autres devoirs de vigilance, mentionnés à l'article L. 1264-1

le prononcé d'une sanction administrative, au terme d'une procédure respectueuse des droits de la défense et du contradictoire. Cet aspect a déjà été intégré au dispositif. Je rappelle aussi que le nouveau dispositif d'interdiction d'activité avant le début de la prestation de l'entreprise étrangère

Cette disposition du code du travail permet à tout salarié étranger qui exerce certaines professions, notamment artistiques, d'exercer son activité en France pendant une durée limitée, sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail. Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d'outre-mer placée sous le régime de l'article 74 de la Constitution. Par conséquent, l'article L. qui prévoit l'obligation de détenir un titre de travail pour les étrangers, sauf en cas de séjour pour motif professionnel de moins de trois mois, ne s'applique pas. L'objectif du Gouvernement est de faciliter les démarches administratives relatives au séjour et au travail sur l'archipel, dans les conditions existant déjà en métropole et dans les départements d'outre-mer. En clair, pour faire la même chose, adoptons un amendement de plus

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à prévoir les modalités de restitution des documents emportés, en cas d'emport de documents lors d'un contrôle en matière de travail détaché.

tant les contrats à durée déterminée sont devenus des contrats de référence au détriment des contrats à durée indéterminée. Ainsi, 87 % des embauches effectuées aujourd'hui le sont en CDD, dont un tiers sont considérées comme très courtes, puisqu'elles ne durent parfois qu'une journée. Pour les autres CDD, plusieurs phénomènes expliquent ce constat : un manque de prévisibilité en matière de santé des entreprises, mais surtout un détournement de la vocation du CDD, dont on fait un outil comptable, soit l'équivalent d'une période d'essai ou d'une période de test. L'enjeu de cet amendement, comme du suivant, est de développer des outils permettant de lutter efficacement contre la recrudescence des contrats précaires, circonscrits dans un temps limité ou à temps partiel. convient de favoriser les recrutements en CDD à temps complet et non à temps partiel, étant entendu que cela coûtera moins cher aux entreprises en fin de contrat, ce qui n'est pas inintéressant. Au premier rang des bénéficiaires de ce dispositif se trouveront les femmes en effet, ces dernières représentent presque 80 % des contrats à temps partiel, plus d'un tiers d'entre elles déclarant vouloir travailler plus. Outre la précarité à l'instant que cela implique, il faut garder en tête que ces pratiques grèvent profondément les conditions conditions de vie des femmes, tout au long de leur carrière et de leur vie, remettant notamment en cause leur droit au chômage et à la retraite. En définitive, un tiers des travailleuses sont à temps partiel, contre seulement 7 % des travailleurs.

CDD. Comme l'a dit mon collègue, 87 % des contrats signés aujourd'hui le sont à durée déterminée. Ce que je veux ajouter, c'est que ce taux a progressé de plus de dix points en moins de vingt ans ! Comme l'a montré la directrice de recherche au CNRS Margaret Maruani, ces contrats sont par ailleurs de plus en plus courts en termes de charge de travail hebdomadaire.

à trouver un temps complet que les hommes. Ces deux freins à l'emploi à temps complet des femmes expliquent aujourd'hui près de 60 % des contrats à temps partiel. De fait, et c'est dans cet esprit que s'inscrit notre amendement, il est urgent de réunir tous les outils existants pour lutter contre le recours abusif au temps partiel, notamment les contrats de très courte durée. Je vous rappelle que le projet de loi relatif à l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, l'ANI, sans revenir sur les critiques que nous avions formulées à l'époque, prévoyait d'instaurer un plancher en matière de contrats à temps partiel, qui était fixé à vingt-quatre heures par semaine. Cette mesure, notre groupe l'a pleinement soutenue, tout en regrettant la multiplication des dérogations.

la loi Travail de 2016 a aggravé la situation en remettant encore en cause la hiérarchie des normes. Comme souvent, il est à craindre que ce ne soit qu'en « tapant dans la caisse si vous me permettez cette expression familière, que nous pourrons sanctuariser ce plancher de vingt-quatre heures hebdomadaires. C'est pourquoi notre amendement prévoit une majoration salariale sur les contrats à faible volume horaire,

contrats à temps partiel, en introduisant une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale. Nous proposons de réduire les allégements de charges sociales sur les bas salaires auxquels ces entreprises peuvent prétendre. Cette disposition, combinée à notre proposition d'instaurer un plafond pour les embauches en CDD, vise à limiter le recours aux contrats courts par les entreprises et, ainsi, à lutter contre la précarité des salariés et, plus particulièrement, celle des femmes. Une étude de la DARES de 2013 a montré que plus de 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Le travail à temps Le travail à temps partiel signifie des salaires, des promotions, des droits sociaux moindres, alors même que l'amplitude horaire et la flexibilité sont bien souvent plus importantes. Or un salarié sur trois déclare ne travailler à temps partiel que faute d'avoir trouvé un emploi à temps plein. C'est ce que l'on appelle le temps partiel subi qui, je le répète, concerne majoritairement des femmes. Dans une optique de recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également de lutte contre la précarité, de manière plus générale, il est nécessaire de limiter ce recours au temps partiel. Dans ce but, nous proposons l'instauration, dans les entreprises d'au moins vingt salariés, d'un plafond d'embauches à temps partiel, fixé à 20 % de l'effectif total de l'entreprise, ainsi que d'une sanction pour les entreprises qui dépasseraient ce plafond.

Cohen, sur l'article. Il est dommage que la discussion sur cet article portant sur l'égalité professionnelle arrive si tardivement, ce qui, je l'espère, n'aura aucune conséquence sur l'approfondissement et la qualité de nos débats.

de rémunération subsiste entre une femme et un homme à contrat, diplôme, expérience et responsabilité identiques. Ce sont les fameux 10,5 % inexpliqués. Avant de passer aux critiques sur les limites de cet article, je tiens tout de même

Comme vous le savez, l'ensemble des organisations syndicales qui ont élaboré une plateforme commune de revendications sur ces questions souhaitent que cet outil soit national, et non à la carte,

Patricia Schillinger. L'article 61 s'inscrit dans le chapitre IV de ce projet de loi et porte plus spécifiquement sur les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes. À travail égal, salaire égal » : nous entendons souvent cette revendication pour plus d'égalité entre femmes et hommes au travail. Malheureusement, nous en sommes encore loin ! En France les écarts de salaires représentent, toutes professions confondues, une différence moyenne de 24 %- en défaveur des femmes, est-il besoin de le préciser

de valeur égale, la rémunération égale entre les femmes et les hommes. En cas de non-respect des indicateurs fixés par décret, les entreprises disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité, sans quoi elles pourront se voir appliquer une pénalité financière. Cet renforce ensuite les obligations des branches en matière de réflexion et d'information sur l'égalité professionnelle, en leur imposant de rendre compte de leur action en matière d'égalité professionnelle dans leur bilan annuel. annuel. Tel est l'esprit de cet article : poser de manière pragmatique les bases d'une meilleure égalité salariale entre femmes et hommes et responsabiliser davantage les acteurs économiques en les amenant à prendre conscience de l'ampleur des enjeux et en les inscrivant dans un cadre contraignant. En le but est de passer, après tant d'années, d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Rossignol, sur l'article. Madame la ministre, je me réjouis que, dans le cadre de ce projet de loi, vous ayez introduit un volet relatif à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Je connais votre engagement sur ce sujet, que je pense à la fois sincère et déterminé. Cependant, je mesure qu'il est difficile d'introduire la régulation qu'exige l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes,

à la fois un enjeu de redistribution des richesses- dans un monde dans lequel la ventilation des richesses entre le capital et le travail s'est profondément dégradée,

aussi d'avoir une palette d'indicateurs permettant de mesurer plus largement l'intégralité de la politique de rémunération et de la progression de carrière. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à réécrire à la marge les articles sur l'égalité salariale, afin de tenir compte de ces évolutions.

Cet amendement vise à rendre automatique la négociation sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. prévoit que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui existe déjà, inclut une négociation sur les mesures de rattrapage salarial. Ce même alinéa prévoit que cette négociation n'a lieu que dans les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale et qui n'ont pas déjà déployé des mesures dans le cadre de la négociation collective. En d'autres termes, les entreprises qui ne sont pas parvenues à l'égalité salariale, mais qui auraient mis en oeuvre des mesures de rattrapage seraient exonérées de l'obligation de négocier. Or il n'existe aucun moyen de contrôler la réalité ni la pertinence des mesures de rattrapage déployées. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être une priorité pour les entreprises. Aujourd'hui encore, des inégalités persistent. En effet, comme tout le monde le sait, les hommes perçoivent en moyenne un salaire supérieur de 22,8 % à celui des femmes, d'après une étude de l'INSEE. Pour cette raison, les mesures de rattrapage salarial devraient faire l'objet d'une négociation automatique dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle. Peu importe que les entreprises aient déjà déployé d'autres mesures, dès lors que l'égalité salariale n'est pas atteinte. L'objectif de cet amendement est de s'assurer qu'aucune entreprise ne bénéficie d'un passe-droit quant à la négociation sur les mesures de rattrapage salarial. Quel

du champ d'application de ce texte. Enfin, je pense que ce sont les plus petites entreprises qui sont les plus exposées aux écarts de rémunération. Dans

vise à renforcer l'article 61 en prévoyant une publicité. Nous voulons en effet nous assurer que les victimes d'inégalités salariales ne prendront pas seulement connaissance du fait qu'elles ont été sous-rémunérées lorsqu'elles seront convoquées chez le DRH et qu'on leur proposera une enveloppe de rattrapage salarial.

Mme Monique Lubin. Lors de sa candidature à un marché public, l'entreprise doit transmettre en annexe le dernier accord relatif à l'égalité professionnelle et la dernière mesure des écarts de rémunération. De cette manière, le pouvoir adjudicateur pourra juger sur place et sur pièces d'éventuels manquements à l'égalité professionnelle et, le cas échéant, avoir connaissance des dispositions prises par l'entreprise pour les corriger. Cette disposition aide également tant les établissements publics que les entreprises candidates à ne pas se placer dans une situation d'illégalité si les secondes remportent le marché proposé par les premiers, alors même qu'elles n'avaient pas le droit d'être candidates. d'augmenter l'effectivité, actuellement peu contrôlée, de l'interdiction de candidater aux marchés publics en cas de non-respect des obligations relatives à l'égalité professionnelle prévue par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.